l'évolution des effectifs, qui reprend un parcours plus réaliste, avec la suppression de 1 850 équivalents temps plein,

d'achever le dédoublement des CP et des CE1 dans les zones REP et REP+. C'est une excellente formule. C'est aussi un effort significatif sur le plan financier. J'ai noté que la dépense représentait 500 millions d'euros pour 300 000 élèves, soit 1 666 euros par élève. L'État investit donc dans la jeunesse française et dans la jeunesse la moins favorisée.

les établissements et qui engage une réforme en amont. Je suis persuadé que vous nous en parlerez. Vous avez opté pour un moyen nouveau : la deuxième heure supplémentaire

L'avantage c'est la sincérité ; l'inconvénient, c'est la soutenabilité dans le temps de votre budget au regard de la loi de programmation des finances publiques.

stable. Les crédits connaissent en effet une hausse modérée, qui s'élève à 1,7 % pour les crédits des cinq programmes de la mission « Enseignement scolaire » qui relèvent de l'éducation nationale, et qui procède essentiellement de l'augmentation des dépenses de personnel et de celles en faveur du handicap. 1 800 emplois, ce qui est faible au regard du plafond d'emplois, qui dépasse le million d'équivalents temps plein. Monsieur le ministre, votre budget est la traduction, certes incomplète, d'une politique dont nous partageons les orientations principales, tout en émettant cependant quelques réserves. Il donne une priorité forte à l'école primaire, dans laquelle notre pays continue à sous-investir, en y poursuivant les créations de postes. Il érige la maîtrise des fondamentaux dès le primaire et la résorption de l'échec scolaire en priorité absolue. Nous ne sommes pas opposés au dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, mais nous vous alertons sur la nécessité d'évaluer rigoureusement cette politique et de faire en sorte qu'elle ne se fasse pas au détriment de la ruralité. Ce sera le sens de l'amendement 2019 verra la mise en oeuvre de la réforme du lycée général et technologique et de la voie professionnelle, où les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements consentis. Nous serons vigilants à ce que cette mise en oeuvre soit à la hauteur des ambitions et qu'elle ne se traduise pas par un accroissement des inégalités entre les territoires. Un chantier demeure, celui de la gestion des ressources humaines du ministère. Avoir des enseignants mieux formés, mieux rémunérés, affectés là où ils sont les plus utiles et dont les obligations de service correspondent à la réalité des besoins, voilà l'enjeu majeur de notre système éducatif ! Il faut donc davantage d'autonomie pour les chefs d'établissement.

Je conclurai en évoquant la scolarisation des enfants de moins de trois ans, sur laquelle j'ai souhaité porter un éclairage particulier. La relance de l'accueil des enfants de deux ans à l'école maternelle, qui était l'une des priorités de la prétendue « refondation de l'école », présente un bilan mitigé, illustrant bien certains écueils de l'action de votre ministère, dont, je vous le concède, avez hérités : absence d'évaluation de ce dispositif, alors que les différentes études réalisées sur ce sujet sont peu concluantes ; dialogue insuffisant avec les communes, acteurs majeurs de cette politique- il est vrai que celles-ci subissent, en même temps, à la fois la baisse des dotations et la réforme des rythmes scolaires - ; absence de priorité clairement donnée aux publics cibles et aux classes dédiées. les enseignants sont peu formés à l'accueil des enfants de cet âge et la formation des ATSEM n'est pas à la hauteur de leur rôle éducatif. Ce sujet met en lumière la nécessité d'un renforcement général de la qualité de notre école maternelle, qui se caractérise par les taux d'encadrement les plus faibles d'Europe et une place quasi inexistante dans la formation initiale des professeurs des écoles.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget de l'enseignement agricole pour 2019 est globalement stable, dans un contexte de baisse des effectifs d'élèves et de nombreuses réformes de fond. Il prévoit la suppression de 50 emplois. Cette réduction, parallèle à celle constatée dans le second degré de l'éducation nationale, est relativement minime, surtout au regard de la baisse continue des effectifs d'élèves et des faibles effectifs par classe. L'augmentation des crédits provient essentiellement des dépenses de personnel, finançant la mise en oeuvre du protocole PPCR et diverses mesures de revalorisation, ainsi que des dépenses en faveur de la prise en charge des élèves en situation de handicap. Ce budget traduit également l'accord conclu avec les familles de l'enseignement privé pour leur financement, qui se traduit par une augmentation de près de 8 millions d'euros des subventions en leur faveur. Accueillant 60 % environ des élèves, les établissements privés sont une composante essentielle de l'enseignement agricole,

comme beaucoup d'entre vous, je crois fortement en l'avenir de l'enseignement agricole. Il répond aux enjeux majeurs que sont la préservation de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, la transition agroécologique et les nouvelles formes d'agriculture. Il constitue également un un levier incontournable pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire, surtout dans les territoires d'outre-mer. Pourtant, l'enseignement agricole connaît une baisse régulière, lente mais certaine, de ses effectifs d'élèves. Celle-ci se poursuit encore à la rentrée de 2018, puisque les effectifs devraient passer sous la barre des 160 000 élèves. Les raisons de cette baisse sont connues : l'implantation traditionnelle de l'enseignement agricole dans des régions en baisse démographique et,, une sous-représentation dans les régions où la demande existe dans certaines régions, une forme de concurrence entre l'éducation nationale et l'enseignement agricole ; surtout, un défaut de notoriété auprès des jeunes. Combien de collégiens savent que l'on peut devenir ingénieur en intégrant une classe de première technologique agricole ? Combien savent que, sept mois après sa sortie de formation, un élève de terminale professionnelle agricole a 59 % de chance de trouver un emploi, contre 42 % pour son homologue de l'éducation nationale ? L'année dernière, je vous disais mon sentiment que l'enseignement agricole devait sortir d'une logique de conservation et de repli pour entrer dans une logique d'expansion. Je me réjouis de constater que le nouveau ministre de l'agriculture, notre ancien collègue Didier Guillaume, partage pleinement cette orientation et cette ambition. L'année 2019 sera déterminante. Elle verra la mise en oeuvre de nombreuses réformes- baccalauréat général et technologique, voie professionnelle, apprentissage -, pour lesquelles l'enseignement agricole a servi de modèle. La coopération avec l'éducation nationale est donc essentielle. Les défis sont nombreux, mais je suis confiant dans la capacité de l'enseignement agricole à les relever grâce à son esprit d'innovation, à la qualité de ses formations et à sa faculté de répondre aux besoins des entreprises et des territoires. Mes chers Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

l'éducation est le premier pilier de la République. C'est un enjeu fondamental de cohésion sociale et de formation citoyenne. Il est donc important que le budget que nous y consacrons soit à la hauteur des enjeux. Cette année, le budget de l'enseignement scolaire augmente modestement, tout en opérant une réduction des emplois. L'examen de l'évolution des crédits rend compte d'une priorité forte accordée par le Gouvernement à l'école primaire, que nous ne pouvons que saluer tant la maîtrise des fondamentaux est primordiale pour l'avenir des 12,8 millions d'élèves scolarisés en France : près de 7 millions dans le premier degré, près de 6 millions dans le second, sans oublier les 260 000 apprentis. Pour prendre en charge ces élèves, pas moins de 881 000 enseignants sont mobilisés chaque année, tous secteurs confondus, dans le système scolaire, constitué de 62 200 établissements. Monsieur le ministre, nous avons la chance d'avoir en France un système éducatif solide mais devenu inadapté, et les études publiées sur le niveau des écoliers français le confirment d'année en année. Malgré les lois qui se sont succédé, le système éducatif français accuse les effets d'une lente dégradation échec scolaire, baisse du niveau de performance des élèves, notamment en français et en mathématiques. Autre fait marquant révélé par le classement PISA : l'école française apparaît comme la plus inégalitaire des pays développés. 73 % des personnes ayant des parents diplômés du supérieur sont elles-mêmes diplômées, tandis que cette part chute à 17 % pour les adultes issus de familles non diplômées. Nous nous situons loin derrière le Canada, la Suède ou la Finlande. Dans son récent rapport publié en octobre 2018, la Cour des comptes constate que l'éducation prioritaire n'a pas atteint son objectif, qui était de réduire les écarts de niveau entre élèves de l'éducation prioritaire et ceux du parcours classique. Ce même rapport établit que les premières années d'étude sont primordiales pour compenser cette perte de chance. Aussi, nous saluons la priorité que vous avez souhaité donner à la scolarisation précoce des enfants, qui reste, malgré les efforts entrepris, en deçà des objectifs fixés à 30 % des enfants de deux ans en REP et 50 % en REP+. L'abaissement de la scolarité obligatoire de six à trois ans va dans le bon sens. Cependant, dans un contexte financier dégradé pour les finances locales, il nous faut veiller à accompagner les communes qui rencontrent des difficultés à dégager les moyens nécessaires à l'accueil de ces enfants supplémentaires. Par ailleurs, la formation initiale des enseignants devrait inclure un module spécifique sur l'accueil de ces très jeunes recrues. Enfin, il appartient au Gouvernement d'évaluer les effets de cette réforme sur la réussite des élèves. Autre mesure phare : le dédoublement des classes de CP et de CE1 à 12 élèves dans les quartiers défavorisés se poursuit, pour s'étendre dès la rentrée de 2019 à l'ensemble des classes concernées. Si notre groupe encourage le déploiement d'un tel dispositif de justice sociale, les collectivités locales sont prises de court, à budget constant, voire en diminution, pour trouver les fonds nécessaires au dédoublement des classes. classes. Nous constatons également dans nos départements que les fermetures de classes en milieu rural restent très mal vécues par les populations locales, qui les ressentent comme un abandon de l'État. Nous sommes donc favorables à l'amendement de la commission de la culture visant à pallier ces fermetures, tout en proposant un amendement de repli que nous vous présenterons. L'attractivité de l'enseignement agricole est un autre sujet fondamental pour l'avenir de nos territoires ruraux. L'érosion des effectifs se poursuit, et cela malgré un bon niveau d'insertion des anciens élèves issus de ces formations. Nous comptons sur l'action du Gouvernement pour valoriser l'enseignement technique agricole, car il se situe au coeur du changement qui anime notre agriculture et nos territoires.

qui rejettent autant votre vision de l'éducation que la politique injuste et méprisante du Gouvernement. Les choix budgétaires que nous examinons aujourd'hui sont incriminés, et il serait bon, me semble-t-il, d'accorder à cette mobilisation toute l'attention qu'elle mérite. Cela serait plus pertinent que d'aviver les tensions, comme à Ivry-sur-Seine, où des lycéens voient leur garde à vue prolongée pour avoir tagué devant leur lycée « Macron démission », ou, ailleurs encore, où l'on répond à des adolescents de seize ans

Les suppressions de postes suscitent colère et inquiétude, comme les réformes qui risquent d'accentuer les inégalités sociales. Votre politique est construite sur ce postulat : la France investirait trop dans le secondaire et pas assez dans le primaire. Ce parti pris vous a conduit à dédoubler les classes en CP et en CE1 en REP et REP+. Mais l'augmentation du nombre de postes n'a pas suivi. Du coup, cette mesure, pourtant louable, s'est traduite par des retraits de postes et donc des classes surchargées dans beaucoup de territoires. Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » a été réduit d'un tiers en 2018 et va continuer à diminuer en 2019. Vous avez justifié cette décision en avançant qu'il n'existait pas de preuves tangibles et scientifiques qu'un taux d'encadrement plus élevé favorisait la réussite. argumentaire est à géométrie variable ! La réduction du nombre d'élèves par classe est la première des priorités pour le CP, mais, « en même temps », on réduit le nombre d'enseignants dans le secondaire et on ferme même des classes rurales au prétexte que le nombre d'élèves y est trop faible. On cherche la cohérence Le jeu de vases communicants auquel vous vous êtes livré pour mettre en place le dédoublement des classes de CP et CE1 pose deux problèmes majeurs. Il est vrai que le primaire est le parent pauvre de l'école française, mais il est faux de croire que le secondaire dispose de moyens suffisants, à plus forte raison au collège ou dans l'enseignement professionnel. Permettez-moi de rappeler que, en vingt ans, la part des dépenses d'éducation a baissé de 1 point de PIB, ce qui représente tout de même 23 milliards C'est d'autant plus problématique que la réforme du baccalauréat demandera un investissement supplémentaire aux enseignants de lycée, dorénavant chargés d'organiser des épreuves et de gérer la place accrue du contrôle continu. Surtout, ces réductions de moyens et d'effectifs sont incompréhensibles au vu des évolutions démographiques. Ainsi, dans le seul secondaire, ce sont plus de 40 000 nouveaux élèves qui sont attendus d'ici à 2021. Au regard de ce constat, vous augmentez les heures supplémentaires des enseignants. Or, d'une part, un enseignant français travaille devant les élèves 900 heures, contre 784 en moyenne dans l'OCDE, et, d'autre part, les équipes éducatives ne cessent de demander des temps hors cours pour travailler sur la vie scolaire et la cohésion au sein du lycée, notamment pour lutter contre les incivilités ou les violences. Face à la crise de recrutement que nous connaissons, ce sont les salaires des enseignants, particulièrement bas en France, qu'il faut augmenter, plutôt que de passer par le subterfuge des heures supplémentaires. Il n'aura échappé à personne, ces jours-ci, que la question du pouvoir d'achat s'impose ... Il serait temps d'y répondre réellement ! Je serai plus nuancée que vous ne l'êtes, monsieur le ministre, sur la hausse de 850 millions d'euros de votre budget

alors que nous approchons des vacances de Noël. Vous savez que ce sujet me tient particulièrement à coeur. D'ordinaire, les situations sont pratiquement toutes réglées entre la rentrée de septembre et celle de la Toussaint.

la voie professionnelle, vous considérez que le lycée professionnel est celui qui « coûte le plus cher et a le plus d'heures de cours sans être synonyme de réussite ». Vous prévoyez la diminution du nombre d'heures d'enseignement. Cela se vérifie, notamment, notamment, à travers l'effondrement des postes de professeurs de lycée professionnel mis au concours pour 2019. Je rappelle que la voie professionnelle est celle qui prépare le mieux les jeunes à l'obtention d'une qualification et à l'insertion professionnelle. Elle permet à de nombreux jeunes, notamment des milieux populaires, d'accéder au bac, puis à l'enseignement supérieur. Elle est également indispensable pour maintenir et développer des savoir-faire, dans l'industrie par exemple. L'apprentissage ne peut pas être la seule réponse, d'autant que la réforme qui dessaisit les régions de cette mission pour la confier aux branches professionnelles risque de porter un coup fatal à de nombreux centres de formation des apprentis, qui maillent nos territoires, et de mener à l'abandon d'un certain nombre de formations.

regroupe l'ensemble des crédits consacrés à l'enseignement scolaire qui relèvent du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Avec plus de 72,762 milliards de crédits de paiement prévus dans le projet de loi de finances pour 2019, la mission « Enseignement scolaire », qui est par ailleurs l'une des plus importantes missions du budget général de l'État, verra ses crédits augmenter d'environ 1,2 milliard hausse de 1,6 % hors inflation. Cette hausse est toutefois moindre que celle constatée au cours du quinquennat précédent, qui s'élevait à 2,4 % en moyenne annuelle.

tous en augmentation, sauf le programme 214, « Soutien de la politique de l'éducation nationale », et en un programme du ministère de l'agriculture, « Enseignement technique agricole », doté de 1,46 milliard d'euros, soit en hausse de 1,4 %. Hors contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions

Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que ces 811 millions d'euros supplémentaires permettront d'être en « capacité d'augmenter le pouvoir d'achat des professeurs ». Cela veut-il dire que cette somme permettra d'honorer la promesse d'octroyer « 1 000 euros de plus à un professeur sur une année en début de carrière » ? Si oui, pourquoi cela n'a-t-il pas été fléché en ce sens dans le bleu budgétaire ? Une telle mesure, découlant des accords « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », décidée par le précédent gouvernement en 2017 et bloquée depuis, est très attendue par le monde enseignant. Contrairement à ce que j'ai pu lire dans les différents rapports et avis sur cette mission, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, son budget se situe donc clairement en deçà des objectifs fixés par la loi de programmation des finances publiques. de finances pour 2019 prévoit la suppression de 2 600 postes d'enseignants, pour 1 900 postes créés dans le premier degré. À ce chiffre s'ajoutent la suppression de 600 postes dans l'enseignement privé et celle de 400 postes administratifs. L'annonce initiale de 1 800 postes supprimés n'est donc pas tout à fait exacte et aura, quoi qu'il en soit, des impacts importants. D'ailleurs, contrairement à ce qu'indiquait le secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, M. Olivier Dussopt, ces coupes ne peuvent pas être justifiées par une baisse des effectifs dans le secondaire, puisque les collégiens et lycéens ne seront pas moins nombreux l'an prochain, bien au contraire ! Il devrait y avoir 40 000 élèves supplémentaires, selon les prévisions de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale, pour chaque rentrée entre 2019 et 2021. Dès lors, la question des effectifs des classes se posera sous peu, ce qui est d'autant plus grave que la France était plutôt bien classée quant au nombre d'élèves par enseignant dans le secondaire.

au collège et au lycée mettra en difficulté certaines académies qui conjuguent faible attractivité du métier de professeur et forte croissance démographique. ailleurs, ces suppressions de postes se marieront mal avec la nouvelle politique publique de réforme du lycée, mise en place dès cette année pour les élèves de seconde pour une expérience sur trois ans, jusqu'au bac 2021. On se dirige, ni plus ni moins, vers une réforme du lycée utilisée comme variable d'ajustement, à moyens constants et avec des postes en moins. Monsieur le ministre, à la lecture de la présentation stratégique de la mission, il semblerait que la première des priorités soit de transmettre les savoirs fondamentaux à tous les élèves et d'agir à la racine de la difficulté scolaire, c'est-à-dire dès les premières années de la scolarité. Vous érigez également la confiance comme ciment de cette ambition : confiance de l'école envers les parents, des professeurs envers leurs élèves, de l'institution envers les professeurs. Vous avez raison. Qui ne partagerait pas cette belle et noble ambition ? Pourtant, et c'est là que le bât blesse, le Gouvernement a-t-il les moyens de ses ambitions ? Se donne-t-il réellement les moyens d'y parvenir ? L'annonce d'une priorité donnée au primaire et d'un maintien des taux d'encadrement dans le second degré, une augmentation imposée des heures supplémentaires sans cotisations sociales, ne va pas dans le sens d'une confiance des personnels dans les orientations de l'exécutif. Je préciserai d'ailleurs sur ce point que les professeurs attendent parfois quatre à six mois pour recevoir le paiement des heures supplémentaires. Est-ce normal ? Le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire- REP et REP renforcé -constitue la principale mesure mise en oeuvre par le Gouvernement en vue de favoriser la réussite à l'école primaire. Mais, pour ce faire, selon les évaluations effectuées par les syndicats et les autres partenaires sociaux, de tels dédoublements consommeraient entre 4 000 et 4 100 postes. À quel niveau seront prélevés les 2 200 à 2 300 postes manquants ? Parmi les 1 496 postes de « maîtres plus » encore existants, ce qui mettrait ainsi fin à cette expérimentation ? Je rappelle que 300 classes ont été fermées à la rentrée de 2018 en milieu rural, du fait du redéploiement des postes pour financer le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire. Assistera-t-on à un de cette mesure pour mener à bien les dédoublements prévus ? Ce n'est pas ce que j'appelle « assurer la continuité du service public sur tout le territoire métropolitain et outre-mer » et faire de l'éducation une priorité ! Je ne m'attarderai pas plus sur ce point, car mon collègue Patrice Joly interviendra spécifiquement sur ce sujet.

ne sont pas non plus acceptables au regard de la situation très difficile que connaissent les services dans ces établissements, déjà fortement impactés par les suppressions successives d'emplois prévues au programme 215. Le redéploiement par transfert

Par ailleurs, il faudra s'assurer que les 1 247 assistants d'éducation seront effectivement présents physiquement dans les établissements. Ils n'étaient que 1 120 selon la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Enfin, si le principal objectif poursuivi par l'éducation nationale, à savoir l'amélioration des performances scolaires, en outre-mer similaire à celui des autres académies françaises, la donne de départ est profondément différente. Il est essentiel que l'égalité réelle outre-mer se concrétise dans le système éducatif, des performances scolaires moindres ne pouvant avoir que des répercussions négatives sur l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et le développement du territoire. L'accès à une éducation de qualité, prenant en compte les spécificités locales pour la réussite et le bien-être de tous les élèves, est également fondamental à ce niveau. Néanmoins, d'importants écarts demeurent du fait d'un décalage persistant entre les ambitions affichées dans les plans d'action, d'une part, et le calibrage des moyens et des besoins, d'autre part. d'autre part. Je prendrai la situation de la Martinique comme exemple : l'affectation massive de nos lauréats hors de l'académie, la diminution importante du vivier des titulaires sur zone de remplacement, quasi vide dans certaines disciplines, et le recrutement de contractuels sur le marché sans aucune expérience sont autant de signes de cette dichotomie. Cela signifie que, chaque année, plusieurs disciplines sont en déficit d'enseignants. Monsieur le ministre, il faut des actes pour garantir que les transformations à venir visent bien des améliorations pour les élèves et les personnels.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous évoquons ce jour les crédits alloués à la mission « Enseignement scolaire », en progression de 1,2 milliard d'euros, soit 1,7 %.

La totalité de cette hausse a vocation à financer des dépenses de personnel, comme des mesures de revalorisation catégorielle, indispensables à une profession dont l'attractivité s'érode année après année. Sur le plan des emplois, 1 800 postes sont supprimés. La priorité demeure à l'enseignement primaire, avec la création de 2 850 postes d'enseignants titulaires. Dans le même temps, 1 050 postes d'enseignants stagiaires y sont supprimés. Sans marges budgétaires supplémentaires significatives, cet effort consenti vers l'apprentissage des fondamentaux se fait aux dépens du secondaire, où 2 650 postes d'enseignants disparaissent, tout comme 550 postes dans l'enseignement privé et 400 postes administratifs. Le principal effort entrepris en direction de l'enseignement primaire continue de résider dans le dispositif de dédoublement des classes de cours préparatoire et de CE1 au sein des écoles situées en réseau d'éducation prioritaire. Nous sommes toutes et tous convaincus du bien-fondé de cette démarche. Lire, écrire, compter, mais également faire preuve de respect vis-à-vis d'autrui sont autant d'éléments essentiels qui nécessitent une attention toute particulière et un apprentissage rigoureux afin d'établir un socle sur lequel tout individu peut ensuite sereinement « construire » son parcours de vie. Toutefois, le dispositif déployé au sein des établissements ne devra pas faire l'économie d'une évaluation prochaine, car sa concrétisation mobilise, au sein du ministère de l'éducation nationale, des moyens importants qui peuvent faire défaut ailleurs. Elle mobilise également des moyens significatifs auprès des collectivités territoriales concernées. Ces dernières, semble-t-il, n'ont pu suffisamment bénéficier des dotations mobilisées à cet effet. Enfin, il apparaît que ces dédoublements de classes au sein des quartiers prioritaires ont « coûté » au monde rural de nombreuses fermetures de classes. Si l'immense majorité des quartiers prioritaires ne se situe pas en zone rurale, ces territoires n'en sont pas moins également en proie à des difficultés sociales importantes. Nous ne le rappellerons jamais assez : une école en zone rurale joue un rôle primordial dans l'attractivité d'une commune. L'accessibilité à une école conditionne bien souvent le départ ou l'arrivée des familles, celles qui, par la suite, assureront le renouvellement générationnel et la vie de la commune. Le groupe du RDSE soutiendra donc l'amendement proposé par notre collègue Françoise Laborde visant à financer la création de 300 postes d'enseignants supplémentaires pour pallier les fermetures observées à la rentrée de 2018 de 300 classes en zone rurale. Notre amendement diffère de celui porté par la commission de la culture, car il ne vient pas ponctionner les crédits dédiés à l'enseignement secondaire, dont les moyens sont déjà amputés dans ce projet de budget. Nous pouvons également observer que ce rééquilibrage salutaire des moyens au bénéfice des écoles primaires est facilité par une dynamique démographique favorable qui conduira l'année prochaine, ainsi que les suivantes, à accueillir un nombre d'élèves décroissant. Toutefois, si le primaire profite d'une conjoncture démographique favorable, il en est tout autrement des établissements du secondaire, qui absorbent actuellement les générations nombreuses du début des années 2000. Il nous faut donc, compte tenu de la baisse des effectifs portée par ce budget, particulièrement vigilants. Ces réductions de postes doivent être compensées par un recours aux heures supplémentaires. Si cette perspective peut être intéressante en matière de pouvoir d'achat des enseignants, elle nous interroge. Initialement tenus d'accepter au moins une heure supplémentaire par semaine, les professeurs ne seront plus en mesure d'en refuser deux si leur établissement leur en fait la demande. Il apparaît toutefois que la moitié des professeurs compte déjà au moins deux heures supplémentaires par semaine. La marge d'augmentation d'heures de cours dispensés ne risque-t-elle pas d'être trop réduite pour parvenir à pallier la baisse des effectifs budgétaires dans le second degré ? J'évoquerai enfin l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire de six à trois ans. Même si sa portée est limitée, avec près de 97 % des enfants de trois ans déjà scolarisés, cette évolution s'inscrit dans le bon sens et continue de recueillir notre soutien. Toutefois, cette nouvelle disposition va engendrer de nouvelles obligations et de nouvelles charges pour nos communes tenues, depuis 1959, de participer au fonctionnement des écoles sous contrat d'association avec l'État. Aucune compensation financière n'est prévue pour le moment dans ce budget. Le projet de loi pour une école de la confiance, présenté ce matin en conseil des ministres, nous apporte des éléments d'information sur l'accompagnement financier dont bénéficieront les collectivités. collectivités. La réponse apportée ne nous apparaît pas satisfaisante, dans la mesure où elle semble reposer sur un principe inédit en matière de décentralisation : quand le Sénat dit « qui décide, paie », le Gouvernement semble répondre « qui faisait quoi avant ? » Monsieur le ministre, toutes les collectivités devront être accompagnées, et pas uniquement celles qui ne le faisaient pas déjà sur la base du volontariat. Je conclurai mon Je conclurai mon propos en évoquant l'enseignement agricole, dont l'attractivité continue de décroître en dépit de la qualité de l'enseignement dispensé et des perspectives d'emplois à l'issue des formations. Nous devons redoubler d'efforts dans la valorisation et la visibilité de ces cursus,

La dernière enquête PISA, publiée par l'OCDE, dresse un tableau alarmant : depuis près de vingt ans, notre système éducatif ne permet plus de réduire les inégalités sociales ni de rendre possible l'élévation des citoyens par le mérite. s'agit pourtant d'un principe cardinal de notre République. Pour relever ces défis, l'école doit se réformer et devenir le socle d'une République avec plus d'égalité, plus de liberté, plus de justice. raison pour laquelle, monsieur le ministre, je souhaiterais, au nom du groupe Union Centriste, saluer la revalorisation du budget de la mission « Enseignement scolaire » avec 811 millions d'euros supplémentaires. Il s'agit d'une réelle source de satisfaction, car ce choix politique sera porteur d'effets concrets sur l'enseignement scolaire. Ce choix renferme également une dimension symbolique forte. En effet, faire de l'enseignement scolaire le premier budget de l'État, c'est envoyer un message clair à nos concitoyens, celui de la priorité donnée au savoir et à la jeunesse. Aujourd'hui, les experts s'accordent à dire que l'État n'investit pas suffisamment, particulièrement dans les premiers niveaux d'éducation. Par ailleurs, toutes les études convergent pour montrer que les inégalités naissent dès l'école maternelle. Pendant trop longtemps, l'école primaire a été le parent pauvre du budget dédié à l'enseignement, inférieur de 14 % à la moyenne de l'OCDE. C'est pourquoi, monsieur le ministre, donner, comme vous le faites, la priorité au premier degré, c'est faire le choix d'une société plus égalitaire. Ce changement de référentiel est donc une bonne chose. Celui-ci passe bien entendu par la transmission et la consolidation des savoirs fondamentaux- lire, écrire, compter -, mais aussi par le respect des valeurs de la République, du principe de laïcité et de l'autorité du professeur. Ce changement passe également par une réorganisation profonde des classes. À cet égard, nous saluons les mesures visant à réduire à 12 élèves l'effectif des classes de CP et de CE1, ainsi que le dédoublement de ces mêmes classes en REP et REP+. Il faudra toutefois veiller à adapter ce dispositif aux écoles situées en milieu rural afin de ne pas accroître la fracture territoriale dont souffrent nos campagnes. Je rejoins, à ce titre, la proposition du rapporteur pour avis Jacques Grosperrin visant à transférer 10 millions d'euros de dépenses du titre 2 vers l'enseignement primaire afin de créer des postes supplémentaires en faveur de l'école rurale. Quant au second degré, nous nous interrogeons sur les suppressions de postes et leur compensation par des heures supplémentaires. Si cette mesure doit permettre d'augmenter le pouvoir d'achat des professeurs, elle reçoit un accueil contrasté de la part des équipes pédagogiques. Le groupe Union Centriste se félicite par ailleurs de l'augmentation des crédits consacrés à l'accompagnement des enfants en situation de handicap, ce qui devrait notamment permettre le recrutement de 1 500 AESH dès janvier 2019. Je souhaiterais conclure en évoquant un sujet qui me tient particulièrement à coeur, celui du harcèlement à l'école. Selon une enquête publiée par l'UNICEF le mois dernier, un tiers des enfants interrogés déclare subir régulièrement des attaques verbales ou physiques de la part d'autres enfants au sein de leur établissement scolaire et 47 % d'entre eux en feraient l'expérience dès le CP. le CP. À l'heure où nous mettons l'accent sur l'importance de l'acquisition des fondamentaux dès le plus jeune âge, il me semble important de rappeler ces chiffres effarants. Des chiffres qui doivent nous amener à réfléchir sur la mise en place de structures d'accueil au sein des établissements scolaires. Car l'enseignement suppose un préalable : la sérénité et la sécurité de nos enfants dans les apprentissages ! Monsieur le ministre, vous l'aurez compris,

M. Max Brisson. Monsieur le ministre, depuis que vous occupez le fauteuil de Jules Ferry, le coeur de votre politique est le dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone d'éducation prioritaire. C'est une bonne décision, je la salue. Elle aura très certainement des conséquences positives sur les apprentissages fondamentaux. Mais cette orientation a d'autres conséquences plus préoccupantes, sur lesquelles je tiens à vous alerter. En zone rurale, la fermeture accélérée des classes et le regroupement à marche forcée des écoles sont contraires aux intérêts des enfants. Élu d'un département de montagne, je peux en témoigner. L'amendement du rapporteur pour avis Jacques Grosperrin souligne l'acuité de cette question. Au-delà, c'est la manière dont l'école replace l'équité territoriale au coeur de ses priorités qui est posée. Autre conséquence du dispositif de dédoublement : la règle tacite du « 80-20 » dans la répartition des moyens entre public et privé n'est plus respectée. L'enseignement privé est soumis bien au-delà des 20 % aux retraits d'emplois, alors que la demande des familles en sa faveur continue de croître. Un tel écart a une cause : la création des postes s'effectue pour l'essentiel en zone d'éducation prioritaire, dont l'enseignement privé est exclu. Résultat : la règle des 80-20 s'applique bien sur les retraits, mais pas sur les dotations, et la balance tacite qui prévaut depuis 1992 n'est plus respectée. Certes, cela pourra évoluer avec les travaux de la mission Azéma-Mathiot et la prise en compte, dans ces dispositifs, des établissements privés qui accueillent déjà en nombre important des jeunes qui relèveraient de l'éducation prioritaire s'ils étaient scolarisés à l'école publique. En attendant, comme vous vous y étiez engagé, on aurait pu espérer une dotation en heures supplémentaires suffisante pour maintenir le potentiel d'enseignement. Or la compensation semble partielle. Il y a donc rupture d'équilibre. d'équilibre. En examinant vos priorités, j'aurais également pu vous parler de la scolarisation des enfants de trois ans, mais je laisse le soin à mon collègue Stéphane Piednoir d'aborder Pour ma part, je tiens à revenir sur la réforme du baccalauréat, autre marqueur de votre politique. Elle comporte des dimensions intéressantes : la suppression des séries de la voie générale, qui devrait mettre un terme à l'hégémonie de la série S l'introduction du contrôle continu, à trop faible dose à mon goût ; la réduction du nombre d'épreuves terminales ; la rénovation de la voie professionnelle visant à regrouper les familles de métiers. Sur tous ces sujets, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire mes espérances et mes inquiétudes. Ces dernières n'ont pas toutes été levées, en particulier sur le bachotage et sur la place de la culture générale dans la voie professionnelle. Or, depuis quelques jours, ces inquiétudes trouvent un nouvel écho, en particulier dans les lycées de la France des périphéries où le désarroi des lycéens rejoint celui des adultes. Aux uns comme aux autres, le Gouvernement doit apporter des réponses. J'ai également eu l'occasion d'appeler votre attention sur les violences subies par les professeurs. Ce matin encore, en commission de l'éducation, l'audition des représentants des syndicats de chefs d'établissement était révélatrice. Au début de nos échanges, ils tenaient avant tout à relativiser les faits avant, finalement, d'aborder la question dans toute sa dimension. Toujours est-il que cela a renforcé ma conviction qu'il est difficile pour les professeurs de se sentir soutenus, tant les personnels de direction- on ne peut totalement les en blâmer -pensent avant tout à défendre l'institution. Pourtant, comme vous le dites souvent, votre ministère est avant tout riche de ses professeurs. Aucune rénovation de notre école ne se fera sans eux. Je veux donc revenir sur les enjeux de la gestion de la ressource humaine, puisqu'elle représente 93 % des crédits de la mission « Enseignement scolaire » et que d'elle dépend la qualité des enseignements. Le mal-être de l'enseignant ne doit pas être sous-estimé. Le combattre est un préalable à toute restauration de l'école de la confiance. Les clés sont connues, nous les avons largement abordées l'été dernier La revalorisation des salaires des jeunes professeurs est la priorité des priorités. Absolument ! Il faut avoir conscience que, dans les grandes métropoles, les jeunes professeurs peuvent parfois s'apparenter à des travailleurs pauvres. La création d'un premier rendez-vous de carrière beaucoup plus tôt est une absolue nécessité. La formation initiale des maîtres doit aussi être remise à plat : place du concours, contenu des formations, rôle de l'éducation nationale employeur, qui ne peut plus être en retenue face aux

à ouvrir ! Le chantier de la formation continue semble tout aussi majeur. Il est paradoxal que le ministère de la formation par excellence soit le plus indigent de tous les ministères quant à la formation de ses personnels. d'une GRH de proximité fait enfin partie de vos priorités, mais elle n'aura de sens qu'avec davantage de personnalisation des parcours et une affectation des moyens qui mette enfin en adéquation les profils des enseignants et les profils des postes, alors que l'indifférenciation des uns et des autres reste la règle commune. Cette GRH de proximité ne sera une réalité que si les rectorats se voient dotés des moyens humains adéquats, ce qui ne pourra se faire que par un effort de déconcentration. Enfin, une GRH de proximité n'aura de réelle existence que si l'on introduit plus de souplesse dans la définition des temps de service à travers leur annualisation et une plus grande présence des enseignants dans des établissements plus autonomes. Plus de souplesse, plus de reconnaissance, plus de formation sont les clés de l'attractivité du métier d'enseignant. Quand ce métier sera redevenu attractif, ce sera le signe que notre école va beaucoup mieux. Je sais la difficulté de lancer de telles réformes. Je connais votre volonté. Je peux apprécier votre discours. Mais je sais ce dont notre école a besoin : ce sont des actes et des décisions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, premier budget de la Nation, d'un montant de 51,7 milliards d'euros et en hausse de 861 millions d'euros, l'enseignement scolaire donne cette année la priorité au premier degré. Lire, écrire, compter, respecter autrui, il s'agit de favoriser, dès le plus jeune âge, la maîtrise de ces savoirs fondamentaux. L'élève pourra ainsi pleinement bénéficier de l'enseignement qui lui sera donné ensuite et développer ses compétences. Pendant plusieurs années, l'effort a été mis sur le secondaire. Cet effort est préservé. Il assure les équilibres primordiaux, tout en mettant l'accent sur la qualité des enseignements, dont le volume est maintenu. La relance des stages de réussite contribuera à l'objectif de réduction des difficultés scolaires. Le dispositif « Devoirs faits » montera en puissance. Pour rendre effective cette ambition d'élever le niveau général, le projet de loi pour une école de la confiance prévoit la scolarisation obligatoire dès trois ans dès trois ans en 2019. Certes, la majorité des enfants de cet âge sont déjà accueillis, mais ceux qui n'ont pas encore accès à l'école sont le plus souvent issus de milieux défavorisés. Or chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, géographique ou culturelle, doit avoir toute sa place à l'école et les mêmes chances de réussite. Dans notre société fragmentée, l'école doit redevenir le premier lieu de justice sociale. Cette réforme ne constituera pas une charge financière supplémentaire pour les communes, car elle sera compensée par l'État. C'est à ce même souci d'équité que répond l'extension du dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire. Là où elle a été expérimentée, les performances moyennes des élèves se sont beaucoup améliorées. Assurer à chacun un véritable droit à l'éducation, c'est aussi veiller à améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap. Des accompagnants seront recrutés. Je reconnais qu'il conviendrait d'améliorer leur statut et leur rémunération. La concertation « Ensemble pour une école inclusive » permettra d'y contribuer. Le lien de confiance avec les membres de la communauté éducative est indispensable à la réussite des élèves. Le caractère attractif du métier d'enseignant doit donc être renforcé, la formation améliorée et la gestion de carrière revalorisée. Vous y travaillez, monsieur le ministre, notamment par un recrutement ciblé, par la mise en place de primes pour les enseignants en réseau d'éducation renforcé et par l'engagement d'augmenter le traitement des jeunes professeurs certifiés de plus de 1 000 euros d'ici à la fin du quinquennat. Toutefois, je crains que Mayotte ne puisse tirer tout le profit de cette politique, tant la situation y est particulière. Elle devrait pourtant en être l'une des premières bénéficiaires. Toute l'île est placée en réseaux d'éducation prioritaire. C'est une bonne initiative, mais le manque de personnels et d'infrastructures en limite la portée. très peu d'enfants de trois ans sont en maternelle. C'est d'autant plus dommageable que le français n'est pas la langue du quotidien. Cela rend difficile l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il faudrait créer une classe par jour. La charge est lourde pour des communes qui ont peu de ressources En 2016, les trois quarts des jeunes de seize à dix-sept ans étaient en situation d'illettrisme, soit sept fois plus que la moyenne nationale. Le nombre d'élèves du secondaire a doublé en dix ans. Par contre, le recrutement des enseignants est difficile et nous manquons de conseillers d'orientation, de médecins et d'infirmiers scolaires. Je me réjouis de la création prochaine d'un rectorat de plein exercice. Sont aussi prévus le recrutement de 500 personnels de l'éducation nationale sur cinq ans et l'engagement par l'État de plus de 500 millions d'euros sur le quinquennat en faveur de l'investissement dans les constructions scolaires. Comment cette ambition se traduit-elle cette année ? Les moyens pour Mayotte sont en hausse, mais certains craignent qu'ils puissent seulement parer au plus urgent, sans impulser un vrai changement de paradigme. Je regrette que, malgré les bonnes volontés et les efforts déployés, notre République ne puisse traiter de façon égale tous ses enfants, fussent-ils à plus de 8 000 kilomètres de Paris. Le groupe La République En Marche votera les crédits de cette mission. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelles doivent être les priorités de l'éducation nationale ? Comment rendre notre système éducatif plus performant, au sens d'une meilleure maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux ? Je suis convaincu qu'il y a, sur ces deux questions, probablement autant d'avis que pour composer l'équipe de France de football à la veille d'une grande compétition internationale. à la première question, monsieur le ministre, vous avez fixé un cap unanimement partagé : lire, écrire, compter, respecter autrui. Ce cap implique que l'on ne dilapide pas le temps des élèves, que l'on se concentre sur l'enseignement de disciplines qui permettront à l'enfant d'acquérir un socle de connaissances indispensables à sa construction et, plus tard, à l'adulte qu'il sera d'avoir des références culturelles solides. J'insiste sur ce point, car j'estime que nous ne pouvons, en période de discussion budgétaire, éluder le sujet du temps d'enseignement nécessaire à l'acquisition de ces savoirs fondamentaux. fondamentaux. Pour prendre un exemple concret, j'estime que le code de la route n'en fait pas partie : l'école ne peut pas, l'école ne doit pas, assurer l'ensemble des missions qui relèvent, pour bon nombre d'entre elles, du cercle familial. Sur la question de l'efficacité de notre système éducatif, nous sommes nombreux à croire que l'essentiel se passe dès l'école primaire. Vous avez fait le choix de porter en grande partie vos efforts sur les dédoublements des classes de CP et de CE1 dans les zones REP et REP+. Je salue bien évidemment cette démarche, qui sera achevée à la rentrée de 2019. il conviendra de faire une évaluation rigoureuse de ce dispositif au regard des quelque 3 900 postes supplémentaires qu'il nécessitera pour sa mise en oeuvre. Raisonner uniquement en termes de moyens est régulièrement pointé comme un prisme réducteur, notamment dans le dernier rapport d'évaluation de la Cour des comptes. Il convient d'y associer une vraie réflexion pour ajuster la gestion des enseignants aux besoins de l'éducation prioritaire. faut-il même imaginer de nouvelles modalités d'affectation et de rémunération des professionnels qui s'engagent sur cette voie. Parallèlement, comme une sorte de corollaire à ces créations d'emplois en zone d'éducation prioritaire, nombre de maires de communes rurales doivent, dans le même temps, faire face à des regroupements, voire à des fermetures de classes. Le climat pesant qui règne aujourd'hui dans notre pays montre combien ces territoires ont le plus grand besoin de politiques publiques efficientes, et pas uniquement en leur faisant jouer le rôle de variable d'ajustement des villes. Les ratios appliqués en zone dense ne peuvent s'appliquer sans discernement aux zones rurales. Pour conclure, je souhaite revenir sur cette annonce du Président de la République relative à l'abaissement de la scolarité obligatoire à trois ans. Cette mesure, qui entrera en vigueur à la rentrée de 2019, n'est pas sans conséquences budgétaires. En effet, si le taux de scolarisation à trois ans est extrêmement élevé- 98,9 % d'après notre rapporteur pour avis Jacques Grosperrin -, il cache des disparités très nettes par exemple, de 70 % à Mayotte. Dans la plupart des communes, on observera une augmentation de quelques unités des effectifs dans les classes, ce qui pourra néanmoins créer quelques surcharges. Mais cette décision entraînera aussi des créations de classes dans un certain nombre de communes, qui devront supporter, la plupart du temps leurs intercommunalités, des investissements importants. Permettez-moi de vous dire que, lors de votre audition du 6 novembre dernier, vous n'avez pas apporté un éclairage très franc sur la prise en charge de ces dépenses supplémentaires. Je sais qu'il devient une habitude de prendre l'argent qui appartient aux collectivités et de ne pas leur donner les moyens d'appliquer les décisions nationales. je m'inquiète de cette nouvelle dépense non compensée, estimée à 100 millions d'euros, et je partage donc totalement la vigilance de notre rapporteur

Comme pour la réforme des rythmes scolaires décidée sous le précédent quinquennat, faire peser ces dépenses sur les collectivités locales sans compensation est profondément injuste. De manière plus conceptuelle, je m'interroge aussi sur la pertinence de cette mesure et sur son éventuel prolongement à la scolarisation des enfants de deux ans. Je suis absolument convaincu qu'il faut respecter le rythme de l'enfant, son autonomie, sa propreté, son aptitude à suivre une journée de classe. Il faut prendre en considération les choix de familles qui considèrent que leur enfant a besoin de plus de temps avant de vivre en collectivité. Cette obligation se traduira aussi par une nécessité de contrôle, qui incombera également aux communes. Je m'inquiète également au sujet des modalités pratiques de la mise en place de cette mesure. Nous le savons bien, lorsque les effectifs le permettent, les plus jeunes sont accueillis de manière très souple dans les très petites sections, pour une intégration progressive au sein de la classe. S'agira-t-il d'une obligation de scolarisation dès trois ans révolus, ce qui signifierait une arrivée de nouveaux enfants tout au long de l'année scolaire, ou bien à l'occasion de la rentrée qui suivra ? de la rentrée qui suivra ? Comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, cette décision soulève nombre d'interrogations que je résumerai ainsi : une même norme, appliquée sans discernement à tous, est-elle cohérente ? Pour tenter un raisonnement par analogie, permettez-moi de prendre l'exemple suivant. Je fais partie de ceux qui pensent qu'une voiture en bon état, circulant par temps clair, sur une route départementale rectiligne et dont le conducteur dispose de toutes ses facultés peut sans risque rouler à 90 kilomètres par heure, À qui viendrait l'idée d'imposer une réglementation plus stricte ? Pourtant, ce gouvernement a fait le choix d'imposer aux automobilistes une décision qui ne tient pas compte de la diversité des routes de notre pays. Rien ne l'oblige à déployer le même rouleau compresseur sur les familles et les enfants, au motif qu'il serait démontré qu'une scolarité anticipée donne de meilleures chances de réussite dans la vie.

Nous ne le rappellerons jamais assez, l'enseignement agricole est et doit rester une filière d'excellence et de réussite qu'il nous faut soutenir.

en hausse ces dernières années, est aujourd'hui stable. Pour autant, nous serons attentifs à la réponse que vous apporterez à notre collègue Élisabeth Doineau sur son amendement relatif à la répartition des 50 postes supprimés, dont 36 postes d'enseignants. C'est en revanche avec satisfaction que nous voyons que les crédits destinés à la prise en charge du handicap atteindraient cette année 3,5 millions d'euros. d'euros. Malgré les efforts budgétaires de ces dernières années, l'enseignement agricole reste encore méconnu. Le nombre d'élèves inscrits dans cette filière est en diminution chaque année, avoisinant les 160 000 pour 2018. Des projets de plans de communication pour mieux faire connaître les spécificités de ce mode d'enseignement, les filières proposées et les méthodes adoptées devaient voir le jour. Est-ce que ce sera pour 2019 ? Nous le souhaitons. Enfin, je voudrais aborder le sujet épineux du nouveau modèle de financement des CFA, qui sera mis en place par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce financement reposera à partir du 1 janvier 2020 sur les OPCO, les opérateurs de compétences, des branches professionnelles. Ce modèle ne correspond pas aux réalités des territoires ruraux,

Le risque à terme est donc de voir disparaître le maillage territorial des CFA. Afin de remédier à ce danger, le Gouvernement nous a annoncé qu'une part du financement serait conservée par les régions pour soutenir les CFA implantés en zone rurale.

sachez, monsieur le ministre, que nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet, afin de nous assurer qu'aucun CFA rural ne ferme à cause d'un manque de financement induit par cette réforme. Pour conclure, j'indique que le groupe Union Centriste votera les crédits affectés à l'enseignement agricole.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission de la culture, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le budget de l'enseignement scolaire qui vous est présenté aujourd'hui traduit la priorité accordée à l'éducation par le Président de la République et le Gouvernement.

Les débats que nous avons ce soir sont à mes yeux significatifs de ce que la démocratie représentative permet de mieux, à savoir la possibilité d'échanger des arguments. Être en désaccord sur certains choix

vous le dis avec une certaine solennité, parce que les prochains jours sont inquiétants. Ce budget approfondit le sillon de la politique lancer l'année dernière. Je remercie les uns et les autres de l'avoir relevé.

Cette priorité me permet d'insister sur l'importance des premiers âges de la vie. Vous l'avez noté, ce projet de loi de finances coïncide avec le projet de loi pour une école de la confiance, que je présenterai en début d'année prochaine et que j'ai présenté aujourd'hui en conseil des ministres.

ans. Cette mesure permettra de faire de la France le pays qui scolarise le plus tôt dans la vie, au moment même où l'ensemble des pays du monde voit, grâce aux progrès des sciences, que les premières années de la vie sont essentielles pour l'acquisition des apprentissages.

je ne me réjouis pas de cette tendance démographique, qui devrait être un sujet de débat très important entre nous. Il y a là quelque chose qui n'est pas sans rapport, selon moi, avec la crise que nous connaissons. À la rentrée prochaine, 2 325 postes devant élèves supplémentaires seront créés dans le primaire

je n'ai pas besoin d'être forcé par quelque événement que ce soit. C'est une conviction que je partage totalement avec vous : nous devons défendre l'école rurale en France, c'est une école qui réussit. Nous devons contribuer à sa renaissance en la plaçant à l'avant-garde des innovations pédagogiques et des éléments d'attractivité. Ne faisons donc pas semblant d'être opposés sur ces questions. Soyons au contraire unis pour arriver au rebond de l'école rurale, dont nous avons besoin, mais qui est rendu plus difficile par les évolutions démographiques dont j'ai parlé. Bien évidemment, ce gouvernement, comme tous les précédents et comme tous ceux qui suivront, tient compte de la démographie. Nous

20 % d'une classe d'âge est concernée par le doublement des classes de CP et de CE1, ce qui coïncide avec les 20 % d'élèves en difficulté pour des raisons sociales dans l'ensemble de la France.

avec l'écart constaté en fin de CP ou en fin de CE1 entre les élèves de certains territoires et les élèves d'autres territoires. Nous devons aussi accompagner les élèves vers la réussite dans le second degré. le volume d'enseignement du second degré public sera-t-il maintenu en 2019. En effet, la diminution de 2 450 moyens d'enseignement, auxquels vous avez fait référence, sera compensée par une augmentation du volume des heures supplémentaires. C'est une mesure qui permettra d'apporter une réponse plus souple aux besoins des établissements. Elle permettra aussi aux professeurs de bénéficier d'une rémunération complémentaire, d'autant que ces heures seront désocialisées. Cette mesure s'inscrit en appui de la politique du pouvoir d'achat, qui constitue un autre pilier de ce projet de loi de finances. Au collège, nous accompagnons plus et mieux tous les élèves vers la réussite. C'est tout le sens de la mesure « Devoirs faits ». Mis en oeuvre à l'automne 2017 dans tous les collèges de France, ce dispositif poursuit sa montée en charge, avec une augmentation de près de 27 millions d'euros

Une augmentation de 4 % des moyens alloués en faveur des bourses de collège et de lycée est prévue. Cela représentera 739 millions d'euros en 2019. En complément, une enveloppe de 65 millions d'euros de fonds sociaux permettra de répondre ponctuellement aux difficultés de certaines familles qui peuvent survenir en cours d'année.

Cette politique nous permet ainsi d'affirmer qu'il y aura toujours un grand nombre d'adultes présents dans les établissements, puisqu'il y aura une assez nette augmentation du nombre d'accompagnants. Les élèves en situation de handicap

à celui des emplois aidés, qui étaient majoritaires jusqu'alors. Ce mouvement se poursuivra en 2019 avec le financement de 12 400 nouveaux emplois d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, dont 6 400 accompagnants supplémentaires au titre de la poursuite du plan de transformation des contrats aidés et 6 000

L'évolution qualitative de l'accueil des élèves handicapés, c'est aussi une évolution de la formation initiale et continue des professeurs, afin que, dans le futur, la formation initiale des professeurs inclue systématiquement cette dimension.

mais c'est aussi la possibilité pour notre système scolaire de prouver que, pour les élèves handicapés comme pour les autres, il est capable de personnaliser les parcours. Dans le

Lors de mon intervention à l'université d'été Ludovia sur l'éducatif numérique, j'ai eu recours à deux mots clés : protection et ambition. La protection répond au besoin d'établir un cadre de confiance. Aujourd'hui même, j'ai signé une convention avec la présidente de la CNIL concernant la protection des données au sein de l'éducation nationale. nationale. À l'issue du discours que j'ai prononcé à la fin du mois d'août, j'ai nommé un responsable national de la protection des données, qui a des correspondants dans chaque académie, pour s'assurer que les données de nos élèves ne servent qu'à leur intérêt et leur éducation et soient protégées des grands opérateurs numériques, qui pourraient en faire d'autres usages. À mes yeux, ce sujet est essentiel. La protection n'est pas une question simplement défensive. Elle est la condition d'une vision offensive du numérique.

domaine. En réalité, plus de 500 millions d'euros sont consacrés à l'innovation, à l'expérimentation et à la transformation de notre système éducatif, au travers du deuxième et troisième programme d'investissements d'avenir, ou PIA, en cours de déploiement. Avec les collectivités locales, nous nous mettons donc en situation d'investir davantage dans le numérique. Enfin, je veux insister sur un point que vous avez été nombreux à aborder, celui de l'attractivité du métier de professeur. Je souligne que le ministère est engagé dans un agenda social depuis le premier semestre de l'année 2018, lequel a vocation à se poursuivre au cours des premiers mois de l'année 2019.

c'est de mieux valoriser l'engagement des professeurs en poursuivant la montée en charge de l'engagement qu'avait pris le Président de la République de relever de 3 000 euros par an les rémunérations des personnels en réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Je vous remercie, monsieur le rapporteur spécial, d'avoir noté qu'il s'agissait d'une évolution très significative. La prime s'est élevée à 1 000 euros à la rentrée de 2018 ; elle sera de 2 000 euros à la rentrée de 2019. Dans le cadre de l'agenda social, nous discutons de ses conditions de mise en oeuvre.

dans notre République -, manifester est un droit, et nous considérons que l'État doit garantir la sécurité de tous, y compris des manifestants. Je ne doute pas que tel sera le cas dans les prochains jours.

privé. Certaines familles scolarisent leurs enfants dans le privé pour des raisons idéologiques, mais c'est assez marginal. Souvent, c'est parce que l'enseignement public ne répond pas à toutes leurs attentes que des familles font le choix d'une scolarisation

agricole. Je ne doute pas que ceux qui en appellent régulièrement à une gestion rigoureuse des deniers publics, et même à une baisse de la dépense publique, auront à coeur, dans ce contexte,

qui ne le sait peut-être pas, que, lorsque Jules Ferry, qui était sénateur des Vosges, donc un Lorrain éminent, a rendu, en 1882, l'instruction obligatoire et gratuite,

raison de le dire. Cette liberté de l'enseignement est donc inhérente à notre culture républicaine et à notre culture nationale. Je ne vois absolument pas la nécessité de la remettre en cause aujourd'hui.

doit respecter une règle de proportionnalité obéissant aussi à une certaine rationalité, surtout lorsqu'il s'agit de mineurs. Je pense, comme vous, je crois, que le surgissement de la violence est un échec collectif, sur lequel il faut que nous nous interrogions. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de renouer, pour l'école,

où de grands syndicalistes d'aujourd'hui ont été éduqués, ouverts au monde et instruits par des congrégations religieuses. Dans cette région, 40 % des élèves sont scolarisés dans des écoles privées,

Aujourd'hui, les villes de Toulouse et de Marseille ont vécu des événements que je considère comme gravissimes et qui sont malheureusement riches de potentialités, elles aussi gravissimes, pour les jours à venir.

pour contrecarrer certaines affirmations. La réforme du baccalauréat est évidemment le résultat d'une consultation extrêmement large : 40 000 lycéens, je le rappelle, y ont participé. Ils l'ont fait notamment au travers d'instances qui sont les plus démocratiques qui soient au sein des lycées, c'est-à-dire les comités de vie lycéenne, qui eux-mêmes se déclinent en comités académiques de vie lycéenne et en un comité national de vie lycéenne. Je suis parfois étonné de voir de toutes petites organisations extrêmement militantes

Je me suis adressé aussi aux élèves, au travers d'une vidéo que chacun peut voir, dans laquelle je leur demande de ne pas aller à ces manifestations, quelle que soit l'opinion qu'ils ont sur quelque sujet que ce soit, parce que, vu les circonstances, ils se mettraient en danger. Je ne dirais pas cela pour n'importe quelle manifestation : ce sont les circonstances

Je vous le concède : l'enseignement privé étant moins présent en éducation prioritaire, un petit changement, de faible nature, est à prévoir. De même, les montants en cause dans les bénéfices que l'enseignement privé peut tirer de l'instruction obligatoire à trois ans ne sont pas grand-chose par rapport à l'évolution d'ensemble que représente ladite instruction obligatoire. Le 80-20

Le budget pour 2019 semble rompre avec cette promesse, puisque ce ministère supportera à lui seul plus de 43 % des suppressions de postes dans la fonction publique de l'État.

de tous les élèves, ce qui implique de doter les enseignants d'une formation initiale et continue de qualité tout au long de leur carrière. Dans ce contexte, il ne paraît pas judicieux de diminuer les crédits qui y sont alloués.

« Enseignement scolaire public du premier degré », afin de financer la création de 300 emplois supplémentaires dans le primaire, compensée par la suppression d'un nombre équivalent d'emplois dans le second degré.

rural. Cette promesse n'a pas été tenue. J'ai bien entendu les propos du ministre, et je connais son honnêteté. Mais fermer une classe en milieu rural- il le sait très bien -, c'est contraindre les enfants et leurs parents à de longs trajets ; c'est programmer

fondamentalement symbolique, permettrait d'envoyer un signal fort en faveur de l'école rurale, à laquelle tous les sénateurs sont attachés et dont le maintien est essentiel à la vitalité et à l'attractivité de nos territoires. Une école qui ferme dans un village, c'est bien sûr le village qui meurt.

! Le RDSE estime que l'enseignement scolaire public du second degré ne peut pas assumer une baisse de 10 millions d'euros supplémentaires de ses crédits. En effet, l'enseignement secondaire subira déjà la perte de 2 650 postes d'enseignants, alors même que 40 000 élèves de plus

nous n'ignorons pas que son action dédiée à la formation des enseignants subit déjà une baisse pour 2019. Toutefois, les parents qui paient pour qu'un enseignement privé soit dispensé à leurs enfants peuvent être

du programme 141 vers le programme 140, afin de financer la création de 150 postes d'enseignants supplémentaires au profit des écoles rurales.

En réalité, l'école rurale bénéficie d'un effort budgétaire sans précédent depuis deux ans. Lors des deux dernières rentrées scolaires, nous aurions dû fermer près de 3 000 classes pour prendre en compte une démographie en baisse de 60 000 élèves

élèves, de 5,5, record historique, contre 5,43 l'année précédente. L'exemple de ce département est généralisable : dans chaque département, le taux d'encadrement s'est amélioré. Je voudrais une nouvelle fois démentir l'idée selon laquelle le dédoublement des classes de CP et de CE1

tous ensemble, notamment pour redonner de l'attractivité aux écoles en milieu rural, au travers par exemple des conventions de ruralité, qui permettent aussi de faire des regroupements d'écoles- on en compte environ 5 000 en 2018. Nous devons aussi prendre en compte les questions périscolaires, avec le plan Mercredi, qui commence à s'appliquer. Par ailleurs- vous y avez fait référence -, la mission « Égalité des territoires », conduite par l'inspectrice Ariane Azéma et par Pierre Mathiot, est chargée de réfléchir à un pilotage vraiment territorial

En application des articles L.O. 151 et L.O. 297 du code électoral, M. le président du Sénat a pris acte de la fin de plein droit, à compter du 5 décembre 2018, à minuit, du mandat de sénateur du Rhône de M. Gérard Collomb. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par M. Gilbert-Luc Devinaz, dont le mandat de sénateur du Rhône commence aujourd'hui, 6 décembre, à zéro heure.

de l'enseignement agricole, qui est victime d'une suppression de 50 postes : une douzaine d'emplois administratifs et techniques, le reste concernant des postes d'enseignants. Parce qu'il est nécessaire de former des jeunes techniciens de haut niveau dans le domaine agricole, notamment au regard des enjeux environnementaux, parce que nous constatons régulièrement que des jeunes sont refusés dans cette voie d'enseignement faute de place, parce que- chacun soutiendra cette idée ici -nous avons besoin de travailler au développement de l'agriculture et d'une agriculture d'avenir,

trouvent souvent un emploi : le taux d'insertion des titulaires d'un diplôme de l'enseignement agricole est supérieur à celui des titulaires d'un diplôme équivalent de l'éducation nationale. Ce sujet me tient

Pendant la même période, les effectifs d'enseignants des trois filières de l'enseignement agricole ont augmenté de 820 postes. En d'autres termes, chaque fois que l'on perd dix élèves, on gagne un poste. Il arrive un moment où il faut se poser des questions. Je pense profondément que les lycées agricoles publics, les lycées agricoles privés, les maisons familiales rurales, par la diversification de leur offre, parce qu'ils proposent à la fois de l'enseignement

tout projet d'effectifs supplémentaires d'enseignants qui s'adossera à une reprise des effectifs d'élèves. Nous ne pouvons pas à la fois défendre l'idée que la dépense publique doit être maîtrisée

Cette diminution continue du nombre de médecins scolaires, experts dans l'exercice de la médecine scolaire, est un frein à la déclinaison de la politique de santé la politique de santé à l'école. Ces médecins détectent des pathologies particulières, notamment chez les enfants et les jeunes de catégories défavorisées. Il s'agit là d'un moyen de détection de ces pathologies irremplaçable.

contre les déterminismes et les inégalités sociales. Ce sont souvent les mêmes enfants qui cumulent les précarités. Je rappelle par ailleurs que l'Académie de médecine

le directeur du service national et de la jeunesse, qui nous a dit avoir constaté que bon nombre de jeunes de seize ans n'avaient pas de carte Vitale, qu'ils avaient des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des problèmes dentaires et qu'ils